madame la présidente,

Après le confinement, après toutes les difficultés, madame la ministre, que nous essayons de juguler avec les plans successifs de relance et de soutien, voilà que l'agitation reprend, le premier jour d'ouverture des magasins,

Elle a entraîné l'annulation des réceptions, événements sportifs et culturels depuis près de huit mois. Du fait du caractère particulier de leurs professions et des outils employés afin de recourir à leurs services, ces professionnels ne peuvent pas bénéficier pleinement des dispositifs de soutien actuellement mis en place par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire dans le cadre du plan d'urgence et du plan de relance. L'assouplissement des restrictions sanitaires à partir de ce week-end ne concerne pas les secteurs ici mentionnés, et les pertes subies en 2020 seront en grande partie irrécupérables. À mesure que la crise se prolonge, que leur activité est maintenue à l'arrêt et que leur situation devient de plus en plus précaire, il apparaît opportun de déployer rapidement un dispositif d'aide pour ces professionnels, afin de répondre à leur détresse. Le présent amendement vise donc à mettre en place et financer un dispositif particulier de soutien à destination des professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel habituellement employés au moyen de contrats à durée déterminée d'usage.

Cela permettrait d'aider ces personnes, qui n'ont plus aucun revenu depuis le début de la crise sanitaire et sont contraintes de recourir au revenu de solidarité active (RSA). Compte tenu des difficultés particulières auxquelles sont également confrontés les professionnels des stations de sports d'hiver, il est proposé de les inclure dans ce dispositif. Pour en assurer la recevabilité financière, l'amendement tend à diminuer de 100 millions d'euros les crédits de l'action n° 01 du programme 305, « Stratégies économiques

d'une part, un renforcement des crédits du fonds de solidarité à hauteur de 1 milliard d'euros pour accompagner l'ensemble des secteurs victimes de la crise ; d'autre part, des mesures de soutien à la relance, avec, notamment, une enveloppe de 400 millions d'euros dédiée à la création de chèques-restaurants pour les ménages les plus modestes.

Vous diminuez les impôts de production de 10 milliards d'euros. Soit, c'est votre choix ! Mais, quand cette réforme prive de 66 millions d'euros la mission d'aménagement du territoire de La Poste, c'est gravissime.

abandonnés par la République. À cet instant, aucun des ministres consultés n'a levé nos inquiétudes. Vous nous dites maintenant qu'une réponse sera apportée en nouvelle lecture. Sachez, madame la ministre, que nous attendons de vous ce soir davantage de précisions,

Il est aujourd'hui essentiel que l'État respecte la parole qu'il a donnée aux élus dans le cadre des contrats de présence postale territoriale. À moins que Mme la ministre, qui semble

sur d'autres continents. À cette fin, le budget de l'AFD devrait être abondé du montant que Proparco pourrait avancer à ces sociétés. Quel est l'avis de la commission ?

Les crédits proposés relèvent donc plutôt d'une logique d'aide au développement, des crédits spécifiques étant d'ores et déjà prévus pour soutenir l'internationalisation de notre économie, notamment le volontariat international en entreprise (VIE), les actions de promotion à l'international ou encore le renforcement des garanties de Bpifrance.

2021. Il doit permettre d'obtenir de nouveaux débouchés pour les entreprises françaises, ce qui nous semble prioritaire. Le débat sur les subventions et prises de participation de l'AFD a, du reste, été tranché hier soir par le Sénat

quelle structure disposons-nous pour permettre aux entreprises françaises d'accompagner leurs partenaires étrangers fragilisés par la crise ? Il n'y en a pas

Ces réformes assurent une simplification pour les entreprises françaises à l'export. Ainsi, ces dernières accéderont plus facilement aux marchés étrangers. À ce jour, la multiplicité des intervenants nous paraît être un frein à l'internationalisation des PME. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la mobilisation des crédits en faveur de l'opérateur Business France. De plus, au titre de la mission « Plan de relance », 100 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus pour financer

est à M. le rapporteur pour avis. Ce deuxième amendement présenté au nom de la commission des affaires économiques vise à doter l'initiative France Num de 5 millions d'euros supplémentaires afin de financer un dispositif de suivi et de mesure des actions de numérisation, ainsi qu'une campagne de communication nationale. Premièrement, France Num ne dispose pas d'un suivi des actions de numérisation engagées grâce à son rôle d'intermédiaire. Il n'a pas même connaissance de leur nombre. Or la politique publique de numérisation des PME, qui s'appuie de plus en plus sur France Num, ne saurait être privée des moyens de suivre et de mesurer l'efficacité de ses dispositifs. Deuxièmement, France Num n'est pas en mesure de connaître sa réelle notoriété au sein du public auquel elle s'adresse, ce qui nuit à l'efficacité de ses outils de communication. les campagnes de communication aujourd'hui menées par France Num empruntent des canaux d'information, dont seuls les dirigeants d'entreprise déjà au fait de l'intérêt du numérique sont familiers. La communication de France Num est donc essentiellement dirigée vers le public qui en a le moins besoin.

portent sur la formation, le conseil juridique, la communication, etc., et couvrent un large champ de domaines : éducation, questions financières, lutte contre l'illectronisme-

également l'occasion de demander au Gouvernement de proposer une stratégie d'ensemble de soutien de l'État aux associations du mouvement consumériste, de réaffirmer leurs missions et d'adapter leurs moyens en conséquence. Sans compenser l'intégralité des pertes cumulées depuis dix ans, cet amendement vise néanmoins à redonner les moyens nécessaires aux CTRC, en revenant au niveau de 2016, soit une hausse de 700 000 euros. Le cycle de consultation et d'accompagnement des associations qui participent au mouvement consumériste a été engagé en février de l'année 2020, dans un contexte- vous l'avez rappelé -de remise à plat des aides aux associations de consommateurs visant à concentrer les crédits sur celles dont le

ces acteurs, qui agissent souvent dans des maisons de la consommation et de l'environnement, sont essentiels face aux profonds changements sociétaux qui touchent le commerce et la manière d'appréhender la consommation. Ces changements mettent en difficulté de nombreuses personnes, souvent les plus fragiles ; la dématérialisation des procédures, l'exploitation des données, tout cela est difficile à appréhender.

mais aussi pour préparer la montée en puissance de dispositifs plus structurants, comme le CyberScore, que nous avons voté il y a quelques semaines et qui va nécessiter une véritable compétence « cyber » au sein de la Les agents de la DGCCRF rattachés au service national des enquêtes (SNE) ont aujourd'hui pour mission de surveiller des secteurs particulièrement concernés par cette fraude. Malheureusement,

sur les services de paiement a renforcé la sécurisation des transactions, notamment des dispositifs de double authentification lors des paiements en ligne. Cependant, un volume important de fraudes à la carte bancaire subsiste et il est essentiel que l'État assume son rôle de protection des consommateurs. De ce point de vue, nous souhaiterions entendre la position de Mme la ministre sur le sujet : les soixante-dix agents affectés à ces missions sont-ils suffisants

ce qui était initialement prévu, précisément parce que le rôle que joue celle-ci dans la lutte contre la fraude, et pas uniquement la fraude à la carte bancaire,

avons revu toutes les participations à des commissions, dans lesquelles leur présence est d'intérêt limité, voire inutile, mais qui leur prenaient du temps administratif qui n'était pas consacré à des missions de contrôle. Cela vaut pour les contrôleurs des directions départementales

afin que sa dotation budgétaire atteigne 1,2 million d'euros en 2021. Le présent projet de loi prévoit en effet que seuls 900 000 euros soient versés par le ministère de l'économie, des finances et de la relance à l'INMA, auxquels s'ajoute une dotation de 600 000 euros versée par le ministère de la culture. Au total, la subvention budgétaire de l'Institut s'établirait donc à 1,5 million d'euros en 2021, contre 1,9 million en 2020. En outre, la dotation devrait n'atteindre que 300 000 euros en 2022, le Gouvernement tablant sur un autofinancement de l'Institut à partir de cette date. Or la crise actuelle entraînera une baisse du mécénat et compliquera la monétisation de ses prestations par l'Institut, rendant peu réaliste l'atteinte de cet objectif d'autofinancement dans les prochaines années. Enfin, certains aspects de l'autofinancement ne sont pas encore expertisés, notamment les risques que ferait peser sur le statut d'association d'utilité publique un assujettissement à la TVA de ses ressources propres.

la gestion du label « Entreprises du patrimoine vivant » pour 300 000 euros, la mission d'observation de veille et d'analyse de l'activité économique et de formation dans le secteur des métiers d'art et du patrimoine vivant pour 250 000 euros, la mission de valorisation des métiers d'art et du patrimoine vivant auprès du grand public en France et à l'international pour 300 000 euros et la mission de de transmission des savoir-faire des métiers d'art et du patrimoine vivant pour 500 000 euros. vivant, développe par ailleurs des ressources propres qui représentent environ 50 % de son budget de fonctionnement pour 2021, grâce à une offre de services

rapporteur spécial. Le présent amendement vise à préserver la ligne prévue pour le financement des activités classiques de garantie de Bpifrance Financement SA sur le programme 134. En effet, pour 2021, l'ensemble des crédits dédiés à ces fonds sera porté par la mission « Plan de relance », et non par des redéploiements internes à Bpifrance Financement SA. Alors que la dotation vise principalement les activités classiques de soutien à la création et à la transmission de petites et moyennes entreprises (PME), il est indispensable de maintenir une ligne dédiée sur le programme 134. L'activité de garantie pour les PME devra en effet être poursuivie bien au-delà de la seule période de la relance, car il ne s'agit pas d'une activité ponctuelle liée à cet le maintien d'une ligne symbolique de 10 000 euros offre aussi l'occasion de dénoncer le financement des activités de garanties par Bpifrance des redéploiements internes, en contradiction avec le principe d'universalité budgétaire. Comme l'indique la Cour des comptes dans son rapport sur Bpifrance de 2016, « ce recyclage constitue une opération de débudgétisation qui prive de fait le Parlement d'exercer son pouvoir en matière budgétaire. Le processus budgétaire normal aurait été celui d'une remontée des dividendes de Bpifrance au budget de l'État et de l'inscription des crédits nécessaires en loi de finances en vertu des principes d'universalité et de non-contraction des dépenses et des recettes.

trace dans le programme 134 de cette mission afin de pouvoir l'accompagner d'une année sur l'autre ; l'avis est donc favorable sur cet amendement.

Cet amendement concerne le respect des règles européennes en matière d'aides d'État. L'article 54 prévoit de prolonger jusqu'à la fin de 2021 le dispositif de prêts participatifs octroyés sur l'enveloppe du Fonds de développement économique et social (FDES) permettant d'accorder des financements subordonnés aux entreprises de moins de cinquante salariés en grande difficulté en raison de la crise actuelle. Nous soutenons entièrement l'initiative du Gouvernement à ce sujet. Cependant, la prorogation prévue à l'article 54 va jusqu'au 31 décembre 2021, alors que le régime temporaire d'encadrement des aides d'État n'est prévu que jusqu'au 30 juin

Préparé avec l'appui de la direction générale du Trésor, cet amendement tend à conditionner le bénéfice des prêts participatifs au respect de ces règles européennes.

qui arrive à échéance au 30 juin, alors que les prêts participatifs sont prolongés jusqu'au 31 décembre.

: La parole est à Mme Évelyne Perrot. Cet amendement de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable vise à compenser les pertes de recettes sur la taxe d'aéroport. Je rappelle que le produit de cette taxe prélevée sur les billets d'avion est reversé aux aéroports pour financer les dépenses de sûreté et de sécurité. La chute du trafic aérien et la perte de recettes de la taxe d'aéroport ont mis en péril ce système de financement. suite aux demandes du Sénat, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 avait prévu le versement d'avances par l'État à hauteur de 300 millions d'euros. Cette enveloppe devrait bénéficier à

L'amendement que je vous présente aujourd'hui vise à accorder une avance de 175 millions d'euros aux aéroports, faute de pouvoir la porter à 350 millions d'euros, en raison de l'insuffisance des crédits disponibles sur le compte spécial pour gager Il s'agit d'une proposition pragmatique et juste ; l'absence d'avance supplémentaire fait aujourd'hui peser un risque de trésorerie majeur pour les plateformes aéroportuaires, particulièrement pour les plus petites d'entre elles. L'État doit prendre ses responsabilités, en assurant le financement d'activités régaliennes qui relèvent de sa compétence.

pour leurs dépenses de sûreté et de sécurité ne sont pas portées par ce compte de concours financiers, mais par le compte de concours financiers « Avances à divers services publics de l'État ou organismes gérant des services publics ». Il y aurait peu de sens à créer deux vecteurs budgétaires pour un seul et même objectif.

d'aéroports frappés par la crise sur le compte de concours financiers « Avances à divers services publics de l'État et organismes gérant des services publics ». D'après les informations dont nous disposons, ce montant est suffisant

: La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier. Cet amendement vise à protéger le financement de l'apprentissage qui constitue une arme considérable dans la lutte contre le chômage des jeunes, sans remettre en question l'objectif d'équilibre budgétaire de France compétences. Le plan de relance ayant pour objectif de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire, il paraît contre-intuitif de conditionner les aides qu'il prévoit à des restrictions budgétaires affectant l'entrée sur le marché du travail d'une génération déjà fortement touchée par la situation actuelle. Il est décisif de continuer à soutenir ces formations, dont les débouchés sont essentiels au fonctionnement de notre pays, comme cela a été mis en exergue par la crise sanitaire. Le PLF prévoit que France compétences prenne toutes les mesures nécessaires pour financer la formation professionnelle continue et l'apprentissage ; or la crainte des acteurs de l'apprentissage est que ces mesures de restriction budgétaire pèsent trop lourdement sur le financement de celui-ci et conduisent des entreprises à fermer des cursus qui deviendraient trop chers et ne seraient pas suffisamment abondés par France compétences. Quel est

effet versé l'année suivant la dépense, alors que la prime est versée de façon contemporaine à la réalisation des travaux, limitant ainsi le reste à charge. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable

Monsieur Meurant,

petites et très petites entreprises de participer à la relance que nous souhaitons tous. La parole est à M.

L'article 56 du projet de loi de finances pour 2021 conditionne l'octroi des aides du plan de relance à de nouvelles obligations en matière environnementale, de parité et de dialogue social. Le durcissement des contreparties demandées aux PME pour bénéficier du plan de relance peut paraître légitime, s'agissant de justifier l'efficience du dispositif de soutien.

: l'organisme chargé de la gestion de l'aide procède à l'examen des dossiers et se réserve le droit de refuser l'octroi d'une aide. Par conséquent, pour éviter les surcoûts et les surcharges de travail pour les PME, mais aussi pour faire en sorte que les entreprises aient un réel intérêt à bénéficier de ces dispositifs, il est demandé, au travers de cet

Une fois les PME exclues, nous avons considéré que l'équilibre auquel étaient parvenus l'Assemblée nationale et le Gouvernement était globalement satisfaisant. En effet, nous considérons que les entreprises de plus de 250 salariés sont capables de réaliser un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre, de respecter des des critères d'évolution des principaux indicateurs de parité et d'informer leurs comités sociaux et économiques.

dupes. Nous ne voterons pas cet amendement de suppression, qui montre que même un peu de conditionnalité, c'est déjà trop pour une partie de la majorité sénatoriale,

Sans précision du caractère direct du bénéfice des aides, la conditionnalité prévue au présent article pourrait s'entendre comme s'appliquant à l'ensemble des entreprises bénéficiaires des garanties octroyées aux fonds de cette mission. La référence au caractère direct du bénéfice doit permettre d'écarter les entreprises bénéficiaires des dispositifs préexistants, qui sont seulement renforcés par la présente mission.

données très basiques ; cela suscitera une prise de conscience collective sans coûter d'argent. Notre objectif est que toute entreprise puisse se livrer à cet exercice sans avoir besoin de faire appel à un consultant extérieur.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises et son décret d'application du 9 août 2017, la France a fait évoluer, sous la forme d'indicateurs

fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. Nous avons déjà un cadre très précis et cet amendement peut faire un lien entre l'aide

de la mission « Plan de relance » à l'application, soit d'une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14 001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système de management environnemental ; soit d'une certification basée sur la norme internationale ISO 50 001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d'énergie par la mise en oeuvre d'un système de management de l'énergie soit d'un label basé sur la norme internationale ISO 26 000 qui propose à tous types d'organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale dans le monde entier. La parole est à M.

Ils demandent simplement aux entreprises qui bénéficient d'un certain nombre d'aides de s'engager dans une démarche pour connaître leur empreinte sociétale et environnementale. Ce n'est rien d'autre que connaître son empreinte, rien de plus

le présent amendement vise à conditionner les aides aux maires au regard des exigences environnementales en lien avec les niveaux E et/ou C de l'expérimentation E+C-environnementale. Ainsi, tous les permis de construire concernant les opérations de logements collectifs, dont la densité est supérieure à un seuil défini ou pour des projets ambitieux, déclencheront le droit à une subvention par mètre carré supplémentaire pour les communes. Quel est l'avis de la commission ? Je peux

problème juridique : le niveau de label n'a pas à être défini dans la loi, puisqu'il relève du domaine réglementaire.

Cette préoccupation apparaît essentielle pour inciter à des constructions sobres en énergie et en carbone, utilisant des matériaux biosourcés et recyclés et respectant la biodiversité.

font ou non le choix de distribuer des dividendes ou de procéder à des rachats d'actions. En tout état de cause, ce qui ne sera pas distribué sous forme de dividendes deviendra une plus-value sur titres,

Le présent amendement vise à formaliser la participation de deux députés du Parlement européen au comité national de suivi du plan de relance.

associer en concertation l'ensemble des parties prenantes à la réussite de la relance- participent à ce comité les organisations représentatives des entreprises et des salariés, les associations d'élus, les parlementaires identifier les pistes d'amélioration et les points de blocage et faciliter et accélérer la levée de ces derniers. Le comité national de suivi a été réuni autour du Premier ministre pour la première fois le 30 octobre dernier.

et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. Deux députés du Parlement européen en sont également membres, mais l'article 56 n'en fait pas mention

... La séance est levée.